aux agents de sécurité privée et aux gestionnaires des sites protégés d'être plus réactifs en cas de menace. La mesure prévue contribuerait également à mieux protéger les sites sensibles contre le risque d'espionnage industriel. Cet article nous permet une nouvelle fois d'observer la dérive que constitue l'évolution des compétences des agents de sécurité privée dans le cadre du « continuum de sécurité », fil rouge de nos interventions. Ces agents ne disposeraient que d'un pouvoir de détection des drones, alors qu'en réalité, en exploitant les informations recueillies, ils sont déjà impliqués dans la procédure de constatation d'une infraction possible, ce qui représente un premier acte d'enquête qui outrepasse, à notre sens, leurs compétences. C'est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.

à neutraliser des drones ni à en actionner eux-mêmes. Ils pourraient simplement les détecter et prévenir les forces de l'ordre, s'ils perçoivent une menace. Il faut certes prendre des précautions, mais on doit tout de même permettre à ces professionnels de s'adapter aux évolutions technologiques, lorsqu'ils exercent leur métier. La

encadre utilement les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée peuvent exercer une activité cynotechnique de prédétection d'explosifs. L'activité privée permet en effet d'accroître le nombre d'équipes susceptibles d'intervenir dans ce domaine, en sus des équipes étatiques. Il semble toutefois nécessaire de tirer pleinement les conséquences de cette mesure, en posant les conditions d'une coordination entre les équipes cynotechniques privées et les services de l'État. Afin de fluidifier l'exercice de l'activité cynotechnique de prédétection d'explosifs, notre amendement tend à organiser un régime de déclaration préalable auprès du préfet. Il est toutefois prévu que cette déclaration s'applique à un lieu et selon une durée donnée, afin qu'une nouvelle déclaration ne soit pas exigée chaque fois que l'intervention d'une équipe est nécessaire. L'amendement vise donc à rendre pleinement opérant l'article 19, sans en complexifier ou en alourdir la mise en oeuvre.

mois. Je crois cependant que, en l'espèce, cette demande d'habilitation est acceptable au regard du caractère technique de la matière traitée et de la nécessité d'avancer rapidement sur ce dossier en prévision des grands événements

par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, est chargé de veiller à l'application des textes en vigueur, et ce dans une démarche partenariale. La composition de ce collège

De plus, ses missions de contrôle et de conseil en font un acteur majeur des relations entre les forces de sécurité et l'État, au vu du développement rapide et des prérogatives sans cesse étendues du secteur privé,

et les conditions d'exercice et de contrôle des activités des organismes de formation dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi. Bien que cet article conduise à mettre le Parlement à l'écart de l'élaboration de dispositions législatives relatives à la qualité et à la fiabilité des formations des agents de sécurité privée, le sujet est d'une nature moins sensible que l'habilitation prévue à l'article 19. Cette Cette habilitation serait justifiée par la nécessité de rationaliser l'offre de formation aux métiers de la sécurité, afin de les professionnaliser davantage, en assurant des enseignements correspondant aux critères attendus et un contrôle homogène de l'évaluation des candidats.

mais qui doivent être encadrés de la manière la plus efficace par l'État qui dispose seul de la compétence régalienne en termes de sécurité. L'État a tenté d'organiser le secteur de la sécurité privée et de contrôler ses agents avec la création du Conseil national des activités privées de sécurité, le Cnaps. Toutefois, comme l'a souligné la Cour des comptes, la création de ce conseil n'a pas permis d'opérer une véritable sélection à l'entrée de la profession ni de l'assainir par des contrôles efficaces. La Cour conclut à la nécessité pour l'État, à tout le moins, d'accroître son rôle au sein du Cnaps en vue d'accentuer les efforts de régulation.

les images des systèmes de vidéosurveillance installés sur la voie publique ou dans des lieux publics. Or le visionnage des images doit être rigoureusement encadré dans le respect des libertés privées et individuelles des citoyennes et des citoyens. Ces garanties impliquent que ces images ne tombent pas entre les mains de n'importe quel agent et ne soient pas utilisées dans n'importe quel but. Aujourd'hui, seuls les agents des services de police ou de gendarmerie peuvent en être destinataires, car ils ont un statut et une formation appropriés à cette prérogative. D'ailleurs, la CNIL n'a pas manqué de rappeler son inquiétude quant à l'élargissement du nombre de personnes pouvant visionner ces images. Les garanties apportées par la commission des lois je suis désolée de le dire, très faibles.. Nous demandons la suppression de cet article afin d'en rester au cadre légal actuel, d'une part, pour ne pas atténuer la frontière entre polices municipale et nationale, car nous estimons qu'elles représentent des entités aux missions et à la composition

Rien dans l'exposé des motifs de la proposition de loi comme dans le rapport de l'Assemblée nationale ne justifie un tel dispositif, qui conduit à ce que les images collectées au moyen de dispositifs de vidéoprotection soient visionnées par un nombre beaucoup plus élevé

autorisés. Ces mesures techniques, dont il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser le détail, permettront une meilleure effectivité des contrôles exercés par la CNIL ou par les commissions départementales. Je veux insister sur l'utilité

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dite Police, justice, a fait naître des dispositions européennes qui devraient s'appliquer à notre droit.

la CNIL ! M. le rapporteur l'a lui-même indiqué : la CNIL relève notamment que les dispositions relatives à la vidéoprotection contenues dans les articles de la proposition de loi « ne permettent [ pas aux responsables de traitement de connaître l'état réel de leurs obligations en la matière ni aux personnes concernées de savoir de quelle manière exercer leurs droits. » On peut donc être contre les caméras de vidéoprotection

et, quand il y a un problème majeur, les caméras transmettent leurs images directement aux tablettes de la police municipale et des gendarmes,

table des mesures qui sont de nature à changer profondément les rapports entre la police et la population.

« déplore qu'une proposition de loi ayant des conséquences aussi graves sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux soit adoptée dans l'urgence, alors que rien ne justifie une telle précipitation

Cela donnait une certaine coloration au débat, chacun se souvenant, notamment ici,

-, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas adapter une loi de 1995, quand bien même elle est le fruit du travail d'un grand sénateur et d'un grand ministre de l'intérieur, l'un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre. Pour ma part, je me félicite de toutes les avancées que le Gouvernement a promues,

! Ces libertés publiques, nous sommes là pour les protéger, je suis d'accord, mais nous sommes également là pour lutter, avec les moyens modernes, contre la délinquance, celle qui embête tous les Français

que le visionnage de ces images doit être rigoureusement encadré, dans le respect des libertés privées et individuelles des citoyennes et des citoyens, et nous refusons que cette possibilité soit donnée aux polices municipales, point barre

amendement a donc pour objet de permettre l'utilisation des images issues des caméras de vidéoprotection pour participer au constat des infractions aux règles de démarchage et de prise en charge illégale de clients par les transporteurs publics particuliers,

Des améliorations ont été intégrées dans la rédaction de l'article 20 par la commission à l'initiative des rapporteurs, notamment en matière de sécurité des enregistrements et de traçabilité de leur consultation. Dans la continuité de ces améliorations, cet amendement a pour objet d'inclure la CNIL parmi les entités consultées avant la prise de ce décret.

traduire les préconisations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour laquelle « il importe que, d'une part, des garanties fortes soient mises en oeuvre pour que seul le personnel dûment habilité puisse effectivement visionner ces images dans le strict besoin de leur mission et que, d'autre part, des mesures de sécurité adéquates soient mises en oeuvre, notamment en matière de traçabilité des accès ». Nous avons évoqué tout à l'heure la nécessité de maintenir

de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Si tant est qu'on puisse l'être, je suis très défavorable à cet amendement du Gouvernement qui entend être habilité à réformer par ordonnance l'ensemble du régime juridique de la vidéoprotection.

c'est de créer les conditions d'une captation d'images dans ces lieux. Pourquoi pas ? ce que je reproche aux auteurs de ces amendements, c'est qu'ils ne vont pas au bout de ce qu'ils pensent vraiment. On nous dit que cela permettrait de diminuer, notamment, les risques de suicide, d'automutilation, d'agression ou d'évasion. Mais il n'y a pas que

au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment, sur présentation de leur carte d'identité professionnelle, les locaux dédiés au visionnage des images provenant de la vidéoprotection. En fait, il s'agit de donner un nouveau droit aux parlementaires, à l'instar de ce qui a été fait par la loi du 15 juin 2000 qui nous donne,

vote. Pour une fois, je suis d'accord avec M. le ministre sur le fait que les parlementaires risquent d'être comme une poule devant un couteau face aux ordinateurs et aux moniteurs

M. Philippe Mouiller. Depuis plusieurs années, nous remarquons la multiplication des systèmes de vidéosurveillance dans les communes françaises : ils ont montré leur efficacité à bien des endroits et dans de nombreuses affaires. Nous sommes nombreux à ressentir une véritable exaspération face aux images de déchets abandonnés en pleine nature, qui, d'une part, gâchent la pureté des paysages, d'autre part, polluent les lieux dans un contexte où le traitement des déchets est une priorité. L'image du maire de Signes, décédé dans l'exercice de ses fonctions, en tentant d'interpeller deux individus en train de déposer illégalement des ordures, est insoutenable pour les élus. Si la loi du 24 juillet 2019 a permis une grande avancée en matière de surveillance à distance de ces dépôts illégaux,

du pouvoir réglementaire. Surtout, comme le Gouvernement l'a rappelé dans sa réponse à une question écrite de Mme Noël, les infractions relatives au dépôt illégal de déchets ne résultent pas de l'usage d'un véhicule : il peut donc y avoir une absence de lien entre l'infraction commise et le véhicule qui apparaît sur l'image.

commission ? Cet amendement vise à rétablir l'article 20 , supprimé par la commission des lois. Nul besoin de préciser que la lutte contre les incivilités urbaines est un enjeu dont les parlementaires,

Si la commission a supprimé l'article 20, c'est que le dispositif voulu par le Gouvernement ne tient pas la route juridiquement. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré en 2010 une disposition qui autorisait la police à accéder aux images de caméras de halls d'immeuble, dès lors que surviennent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de la police ou de la gendarmerie. Le législateur a ensuite revu sa copie et a prévu des garanties jusqu'alors manquantes : premièrement, la transmission des images n'est déclenchée qu'en réponse à un risque caractérisé deuxièmement, elle ne doit durer que le temps de l'intervention de la police. Le Gouvernement, en voulant rétablir l'article 20 , cherche à supprimer toutes ces garanties opérationnelles qui sont à nos yeux indispensables.

disposant que, lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de police ou de gendarmerie ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, le propriétaire, l'exploitant de ces immeubles ou leur représentant peut rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en oeuvre dans les parties communes.

L'article 20 ouvre la faculté de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmis au sein des salles de commandement de l'État aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF. Cette mesure à visée uniquement opérationnelle serait justifiée par la volonté de renforcer la coordination des services de police et de gendarmerie et des services de sécurité internes précités dans la perspective de la création d'un futur centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France. telle disposition conduirait à allonger une fois de plus la liste des personnels habilités à visionner des images et enregistrements de vidéoprotection. qui soulève une difficulté d'application de la mesure au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en raison de la nature privée du statut des agents de sécurité de la RATP et de la SNCF.

on n'imagine pas que, dans l'exercice de leurs missions, il leur soit possible de s'en tenir exclusivement à de la coordination. Or l'exercice des prérogatives de puissance publique est réservé aux seuls agents publics des forces de sécurité. C'est pourquoi le dispositif ne semble pas suffisamment proportionné. Ainsi que le souligne la CNIL, la transmission en temps réel de ces images, en dehors de toute réquisition judiciaire, ne devrait être justifiée que dans des cas précisément définis

complémentaires à ce dispositif. Les agents privés auront vocation à n'être destinataires que des seules images captées sur leurs emprises respectives. La consultation des images aura lieu uniquement sous l'autorité et en présence d'agents des forces de police ou de gendarmerie, avec pour finalité exclusive la coordination des interventions avec lesdites

d'une délégation à des personnes privées d'une mission de surveillance de la voie publique, ce qui est bien entendu contraire à la Constitution. Au regard des enjeux financiers et de sécurité, la commission a fait son possible pour rendre cette

car ces dispositions portent atteinte, à de nombreux égards, à l'exercice des droits et libertés fondamentales comme le respect de la vie privée, mais également la liberté de manifester- ce dernier point concerne spécifiquement les drones. Nous y sommes opposés ensuite du fait de l'utilisation prévue de ces technologies hautement intrusives. En effet, nous estimons que la vocation première des caméras-piétons est d'être un outil de contrôle du comportement de l'agent. Nous regrettons que cette précision n'ait pas été introduite dans le texte. Nous regrettons également qu'aucune disposition ne vienne expliciter leur utilité, notamment lors de procédures à l'encontre de l'agent. Par ailleurs, l'accès qui serait donné à ce dernier aux images limiterait cette capacité de contrôle, en permettant d'adapter les discours aux faits, que le relève la CNCDH. En outre, nous contestons que, dans la pratique, notamment du fait du manque d'autonomie des batteries utilisées par ces caméras, ce soit l'agent lui-même qui déclenche cet outil. On doute qu'il la déclenche en pleine commission d'une infraction ... Enfin, en ce qui concerne les caméras embarquées, des lieux d'habitation ? Quelle protection ce texte prévoit-il ? De manière générale, les garanties sont lacunaires.

Il me semble que l'équilibre trouvé par la commission, qui a ajouté plusieurs précisions au texte, est désormais satisfaisant. Concernant la possibilité de consultation des images lors des interventions, la commission a précisé les conditions opérationnelles justifiant cette consultation immédiate- par exemple, faciliter la recherche d'auteurs d'infraction, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions -et-et ajouté une exigence de traçabilité des consultations ainsi réalisées, pour avoir la garantie que les images ne puissent pas être supprimées sur l'appareil lui-même.

ainsi libellé : La parole est à Mme Esther Benbassa. La vidéosurveillance présente un risque d'atteinte à la vie privée et son utilisation doit donc être strictement nécessaire et proportionnée pour atteindre un objectif légitime. Nous estimons qu'il ne peut pas être laissé trop de latitude à la définition de l'utilisation des caméras individuelles, technologie de contrôle intrusif : si elles doivent être déployées, nous souhaitons à tout le moins y associer des garanties liées au respect du droit à la vie privée. Il apparaît donc essentiel qu'à ces mêmes articles la loi affirme clairement que l'utilisation de ces caméras individuelles a pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences policières. N'oublions pas que l'une des vocations des caméras-piétons est d'être un outil de contrôle du comportement du fonctionnaire de police ou du gendarme. En ce sens, elles représentent un atout dans le contrôle de l'action des agents, notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires dans le cadre d'une mise en cause d'un agent pour une infraction commise pendant l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'encontre d'un agent, ces images devront être transmises sous scellé

de lutter contre les violences policières et d'interdire le couplage des caméras individuelles avec des dispositifs de reconnaissance

Mme Esther Benbassa. Parce qu'ils traitent tous du déploiement et de l'intensification de la vidéosurveillance mouvante, il aurait été utile de traiter les articles 21, 22 et 22 ensemble, puisqu'ils disposent respectivement des caméras-piétons ou caméras individuelles, des caméras aéroportées ou drones et des caméras embarquées. Nous regrettons que la commission des lois, qui a amendé les dispositions de l'article 22 ayant trait aux drones pour y ajouter des garanties relatives à la reconnaissance faciale et au fichage- ce que, bien sûr, nous saluons -, n'ait pas pris la peine d'apporter ces mêmes garanties pour les caméras individuelles. Or, pour celles-ci, ces garanties nous paraissent d'autant

d'interdire l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale et les interconnexions automatisées de données qui peuvent être effectuées lors de l'analyse des images des caméras individuelles. Le recours à cette technique semble devenu systématique, tout en ne reposant sur aucun contrôle du principe de proportionnalité

: La parole est à M. Jean-Yves Roux. L'article 21 vise à faciliter le recours aux caméras mobiles par les agents de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que par ceux de la police municipale. Nous nous réjouissons de la position de la commission des lois et des modifications adoptées à l'initiative de nos rapporteurs. Cela a été souligné, l'usage des vidéos n'a pas une vocation illustrative ni polémique, mais doit servir les agents dans leurs interventions, le maintien de l'ordre et la sécurité de nos concitoyens. Toutefois, une disposition peut paraître étonnante : il est question que, lorsque la sécurité des agents ou celle des biens et des personnes est menacée, les images captées au moyen de caméras individuelles puissent être transmises en temps réel au poste de commandement. Elles le « peuvent », ce n'est donc pas une obligation. Cette transmission devrait justement être obligatoire, et non pas une simple possibilité offerte aux agents intervenants. L'objet de cet amendement est de procéder à une modification en ce sens. Quel est l'avis de

Nous y sommes défavorables, monsieur le président, parce que cet amendement vise à supprimer les remontées d'informations au ministère de l'intérieur concernant l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.

utile, puisqu'il vient combler un vide juridique, en proposant de définir le cadre légal d'utilisation des caméras aéroportées. La nécessité d'inscrire dans notre droit un régime dédié à l'utilisation de cette technologie s'imposait d'autant plus que le Conseil d'État avait pointé une atteinte « grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée » à l'occasion de son utilisation par les forces de sécurité.

lois, comme l'interdiction de la captation des sons, de la reconnaissance faciale et des interconnexions automatisées de données, les garanties censées assurer le respect de la vie privée sont insuffisantes et inappropriées. En effet, l'article 22 ne précise pas comment il sera possible de rendre compatible l'usage des drones avec la condition impérative de ne pas visualiser les images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées. De plus, les modalités de l'information du public ne sont pas précisées, sauf à se satisfaire de la formulation « par tout moyen approprié ». En outre, ces protections sont aléatoires, car elles se trouvent conditionnées par des réserves qui les rendront le plus souvent inapplicables. D'ailleurs, sur ce sujet, la commission des lois n'a pas apporté de réponse. Il n'est pas acceptable que le Parlement ne se prononce pas sur cette condition minimale, en se déchargeant sur le pouvoir réglementaire par un renvoi à un décret d'application. Le périmètre servant de support est trop lâche en raison de la multiplicité et de la diversité des motifs susceptibles d'être invoqués pour justifier le recours aux drones à des fins de captation et d'enregistrement. À cet égard, la mobilisation de caméras aéroportées, notamment pour l'encadrement des manifestations, ne va pas sans soulever de fortes craintes sur le risque d'atteinte au droit de manifester.

particulièrement adaptés : les infractions graves ou les lieux difficiles d'accès ou exposant les agents à des dangers particuliers. Nous souhaitons aussi prévoir un régime souple d'autorisation par le préfet ou le procureur, selon les cas, lorsque les drones